J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur la proposition de loi relative à l'encadrement de l'usage du téléphone portable dans les écoles et les collèges est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

voter pour. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique du scrutin. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

hors continuité comme zone à urbaniser. Le PLU peut aussi délimiter des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ou des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées.

raisons. D'abord, nous ne partageons pas le recours systématique aux ordonnances, notamment quand il s'agit de toucher au code de l'urbanisme, si sensible pour les collectivités territoriales.

aux directives paysagères : autant de documents qui doivent être particulièrement suivis et pour lesquels nous souhaitons que soit maintenue la notion de compatibilité ! Nous sommes également opposés à la suppression de la notion de prise en compte, qui permettait une cohérence globale entre tous les documents d'urbanisme. Sous prétexte de simplifier et de favoriser la construction de logement, l'article 13 déréglemente purement et simplement le droit de l'urbanisme, offrant la possibilité aux documents d'ordre inférieur de s'affranchir des règles nationales.

simplifier la hiérarchie des normes des documents d'urbanisme, hormis dans l'étude d'impact, où il est indiqué : « La technicité des dispositions à modifier et l'exigence de concertation avec les associations de collectivités territoriales justifient le recours à une ordonnance dont l'article d'habilitation Nous le savons, la simplification et la rationalisation de ces documents sont souhaitées par tous les acteurs locaux. Mais la compatibilité entre les normes en matière d'urbanisme est un sujet important ; elle pourrait impliquer des modifications du contenu du SCOT et l'adaptation du schéma Issue d'une procédure longue de débats parlementaires et de concertation avec les acteurs des territoires, cette articulation ne peut pas être modifiée aujourd'hui par la seule main du Gouvernement. Face à l'imprécision du cadre de l'ordonnance, nous saluons les modifications apportées en commission visant à préciser que les obligations de prise en compte pourront être supprimées dans certains cas au profit d'une obligation de compatibilité, mais que cette suppression ne sera pas appliquée de manière uniforme et indiscriminée. Par ailleurs, le Gouvernement se donne un délai de dix-huit mois pour rédiger ces ordonnances. Ce délai sera-t-il suffisant pour organiser la concertation et lever les contraintes opérationnelles des collectivités ?

la qualité et le caractère du patrimoine, la qualité du projet et la capacité de l'organisme de gestion à conduire ce projet. La charte est élaborée par les parcs, les élus, les agents et les partenaires. Elle est soumise à enquête publique. Elle est approuvée par les communes constituant le territoire du parc, par la ou les régions concernées, ainsi que par les partenaires socioprofessionnels et associatifs. Enfin, elle est approuvée par le ministère de l'environnement. Nous ne pouvons pas balayer d'un revers de main les chartes des 53 parcs naturels régionaux, qui représentent 15 % du territoire français, 12 régions, 74 74 départements et 4 400 communes ! Les parcs sont des laboratoires d'idées, d'expérimentation, d'innovation, d'éducation, d'information, de développement économique et social, de protection et de gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager. C'est le coeur de ce projet de loi d'aménagement du territoire.

Par une application locale fine et partagée, les chartes permettent d'inciter fortement les collectivités à intégrer les enjeux de développement et d'aménagement durable, de protéger les patrimoines, les paysages, la biodiversité, de limiter l'artificialisation et la consommation des espaces.

vise à assurer l'opposabilité des chartes des parcs naturels et régionaux aux documents d'urbanisme. Ces chartes sont des documents issus d'une importante concertation locale. Elles garantissent le cadre environnemental, agricole, forestier et paysager de ces lieux de vie et de leurs ressources.

l'avis de la commission ? Lors de l'adoption du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Sénat s'était prononcé en faveur de la sauvegarde d'un rapport de compatibilité entre les documents d'urbanisme et les chartes des parcs naturels régionaux.

? Non, monsieur le président.

explication de vote. Il faut dix ans pour élaborer une charte de parc. Comme élue, j'ai travaillé trois fois dix ans pour le renouvellement de la charte de mon parc.

il s'avère que l'articulation entre ces documents n'est pas optimale. Alors que la loi ALUR a engagé un rapprochement du PLU, du PLH et du PDU, il conviendrait d'aller plus loin et de fusionner ces trois documents de planification et de programmation d'échelle intercommunale.

est ainsi libellé : La parole est à Mme Valérie Létard. Les terrains situés dans les secteurs urbains sont grevés de servitudes et de droits réels institués afin de répondre aux contraintes urbaines du XlX et du début du XX siècles, et alors justifiés par l'existence d'un tissu urbain fortement résidentiel. Au regard des évolutions réglementaires et urbaines, ces servitudes ne paraissent plus adaptées et constituent des freins à l'acquisition de foncier ou à la réalisation d'opérations de construction. En conséquence, il est proposé de compléter l'article 703 du code civil, afin que la disparition totale et irréversible des éléments essentiels à l'origine de la création de la servitude soit une cause d'extinction de celle-ci. Quel est l'avis de la commission ? Si la commission partage l'objectif de rationalisation des servitudes d'urbanisme anciennes, qui limitent les droits à construire, elle se pose la question de l'opportunité de prévoir que la simple délivrance d'une autorisation postérieure rende les servitudes

créées dans l'intérêt général. Comme vous l'indiquez, madame la sénatrice, la disparition totale et irréversible des éléments essentiels qui étaient à l'origine de la création de celles-ci permet la mise en oeuvre des projets d'urbanisme. En l'état actuel du droit, il existe déjà divers mécanismes pour faire prévaloir les règles d'urbanisme sur les règles de droit privé. Pour citer le cas le plus courant, les règles de droit privé des lotissements peuvent être modifiées par les colotis ou par le maire, afin de les mettre en concordance avec le PLU.

M. Jean-Marc Gabouty. L'article L. 442-9 du code de l'urbanisme prévoit que certaines dispositions non réglementaires qui sont contenues dans un cahier des charges d'un lotissement deviennent caduques à compter du 24 mars 2019. Il s'agit des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire, d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble. Toutefois, les colotis peuvent maintenir ces clauses à condition de procéder à la publication du cahier des charges au service de la publicité foncière. La majorité qualifiée des colotis s'applique en ce cas. Pourtant, le droit en vigueur permet aux colotis de modifier les règles internes au lotissement à la majorité qualifiée et à la commune de procéder à la modification des documents du lotissement pour mettre en concordance les règlements et les cahiers des charges avec le PLU. À des fins de simplification et dans l'objectif de garantir le respect du principe de liberté contractuelle, en particulier le droit au maintien des conventions légalement formées, le présent amendement vise à supprimer le dispositif de caducité automatique.

Cet amendement porte sur le dispositif de caducité de certaines clauses de cahiers des charges de lotissements concernant les parties communes. Les nouvelles contraintes en matière d'urbanisation, notamment les exigences de densification, couplées à la nécessaire réhabilitation de certains espaces verts, qui sont nombreux au sein d'anciens lotissements, posent la question de la pertinence du maintien de l'accord unanime des colotis prévu par la loi ALUR. L'accord unanime des colotis devient un frein important pour la commune, qui ne peut plus réaliser ses missions en matière d'aménagement. C'est également, il ne faut pas le négliger, une porte ouverte à des litiges ou à des procédures contentieuses, qui se multiplieront dans les années à venir, au rythme des reconversions d'anciens lotissements. Cet amendement vise donc à assouplir cette règle pour que les parties communes des lotissements soient assujetties aux mêmes règles que les documents du lotissement- règlement, cahier des charges, etc. -en permettant une modification à la majorité qualifiée et non à l'unanimité des colotis. La parole

afin de l'urbaniser. La règle de l'unanimité reste de mise. Or cette différence de régime juridique, selon que la modification concerne ou non les parties communes, ne se justifie pas et entrave la densification de certains lotissements.

que celles qui prévalent au moment de la délivrance du permis d'aménagement du lotissement. Si le PLU évolue par la suite, cela n'aura pas d'effet sur les constructions des lots individuels. Cet amendement va dans le bon sens et permettra de sécuriser les habitations construites en lotissement. Avis favorable.

qui nécessite un maximum d'échanges et un partenariat solide entre tous les élus concernés. Pour parler de la terre qui me concerne, les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais, comme l'aurait si bien dit le docteur Aliker, mort à 106 ans,

Or, à cette date, il est peu probable que la MGP ait, d'une part, adopté son plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, ou PMHH, et donc ses orientations en matière de production et de financement du logement social, et, d'autre part, mis en place les mesures nécessaires à cette prise de compétence.

en créant notamment une discontinuité dans la politique de financement du logement social, risque de retarder les projets de création de logements sociaux et de pénaliser les communes en milieu de période triennale de rattrapage SRU. De plus, alors que les établissements publics territoriaux sont réaffirmés comme échelon de rattachement des offices publics de l'habitat, ils ne seront plus compétents pour financer les opérations de leurs propres offices. Déjà reporté d'un an par la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, le transfert des compétences « financement du logement social » et « aménagement des aires d'accueil aux gens du voyage » vient de nouveau de l'être, avec sagesse, par l'Assemblée nationale, « à la date à laquelle le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est rendu exécutoire ». Toutefois, il paraît indispensable de stabiliser les modalités de financement du logement social,

confier l'exercice des compétences « aides financières au logement social », « actions en faveur du logement social » et « actions en faveur du logement des personnes défavorisées » aux établissements publics territoriaux en lieu et place de la Métropole du Grand Paris. n° 104 rectifié, de repli, tend à reporter le transfert de compétence des territoires à la Métropole du Grand Paris au 1 janvier 2021, date par ailleurs plus cohérente avec d'autres dispositions à venir, notamment les opérations de regroupement des offices d'HLM.

Je tiens à rassurer Christine Lavarde : la Métropole du Grand Paris a délibéré et a adopté son PMHH. Il faut rendre ce dernier exécutoire. Si on a reculé la date initialement prévue, c'est que la Métropole du Grand Paris s'est mise en place le 1 janvier 2016

12 PLH approuvés avant le 31 décembre 2015, mais pas encore exécutoires à cette date. Cela compliquerait la conduite des politiques locales de l'habitat sur le territoire de ces PLH.

de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres. Cet outil puissant permet à cette métropole de s'appuyer sur les compétences de certains services communaux, le temps que cette organisation encore récente devienne pleinement organisée et parfaitement opérationnelle. À l'inverse, les établissements publics territoriaux, les EPT, ne peuvent confier la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement relevant de leurs attributions aux communes membres. Il serait logique qu'un tel mécanisme puisse être mis en place. Quel est l'avis de la commission

Merci, monsieur le ministre,

chers collègues, l'architecte des Bâtiments de France est un fonctionnaire qui travaille dans une unité départementale de l'architecture et du patrimoine, une UDAP, sous l'autorité du préfet de département, lequel le note. Par ailleurs, il appartient aussi à la

mais celle de la mission de service public que les ABF doivent remplir au nom de l'État, au titre de leur compétence en matière de préservation du patrimoine.

Pourquoi ne cite-t-on jamais les cas dans lesquels l'intervention de l'ABF a permis non seulement de protéger un patrimoine historique qui allait être détruit, mais aussi de réduire les coûts d'opération ? Permettez-moi de vous donner un exemple : la réhabilitation du couvent de Kerlaouen, à Landerneau,

pour préserver un patrimoine qui, vous le savez, constitue une part importante de l'âme de notre pays, de nos villes, de nos villages, de nos centres-bourgs et de nos campagnes, et qui participe à la qualité de vie recherchée par nos concitoyens. Ce

Lorsque j'ai un choix à faire, je privilégie l'intelligence territoriale, l'intelligence du maire et du conseil municipal, quel que soit mon respect pour la position de l'administration.

prendront leur décision. À l'arrivée, qui sera souverain ? Le citoyen et l'électeur, lors des prochaines élections municipales ! C'est la raison pour laquelle

Soyez-en sûr, nous garantirons toujours aux ABF le rôle primordial de protection et de conservation de notre patrimoine. Mais, parce que nous faisons confiance aux élus locaux, nous leur accordons deux possibilités de dérogation, bien encadrées, à l'avis conforme de l'ABF. Nous ne prenons pas de risques importants en laissant aux élus locaux, auxquels nous faisons confiance, cette marge de manoeuvre ; nous accélérons les procédures. De plus, en cas de désaccord, le processus de discussion sera simplifié à la saisine d'un médiateur. Cette procédure permet aux acteurs de prendre leurs responsabilités pour tendre vers une solution commune. Lorsqu'il faut détruire un pylône de téléphone aussi vite, voire plus vite, qu'on ne l'a construit, lorsque des familles vivent dans un habitat indigne et insalubre, il est de notre devoir, mes chers collègues, de prendre nos responsabilités et d'éviter toute rigidité et toute lenteur dans la revitalisation de nos territoires. La parole

d'une commission mixte paritaire, à une majorité de deux voix, que cet avis conforme soit maintenu. Moi-même, en tant que maire, je me suis heurté

Seule l'Italie peut rivaliser avec elle, et encore ... Ces trésors que nous ont légués nos pères, qui sont admirés dans le monde entier et attirent des millions de touristes passionnés par l'art,

parce qu'ils aiment leur ville et savent très bien que l'attractivité de leur territoire dépend en grande partie de ce patrimoine. Je suis élu de l'Oise et Beauvaisien.

Je ne connais pas de maires qui souhaitent défigurer, enlaidir, vandaliser leurs quartiers historiques. Les élus locaux ont effectivement comme les associations de sauvegarde du patrimoine- je pense à la Fondation du patrimoine de mon ami Alain Schmitz -, et comme les architectes des Bâtiments de France, dont les conseils avisés donc toujours précieux. Dans le meilleur des mondes,

cette notion d'avis conforme et cette impression de toute-puissance des ABF sont parfois ressenties comme un abus de pouvoir par les élus locaux. Si je fais confiance

par les élus locaux que nous représentons ? Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux : les ABF sont là pour remplir leur rôle, qui leur est confié par l'État ; les élus sont là pour investir et bâtir dans leur territoire, ce qu'ils font très bien. N'affaiblissons ni les uns ni les autres ; maintenons l'avis conforme des ABF. La

sûr ... Comme beaucoup d'entre vous, j'ai une expérience d'élu local- adjoint à l'urbanisme, au logement, président d'agglomération -, et puis, comme beaucoup d'entre vous, j'ai beaucoup circulé dans ce pays,

j'ai rencontré la ministre de la culture et son cabinet, j'ai simplement exprimé ce que j'entends sur le terrain et ce que j'ai constaté dans l'exercice de mon mandat d'élu local.

par rapport aux autres pays, nous avons la chance d'avoir ce patrimoine, cette culture. On ne va pas faire passer le droit au logement avant le droit au patrimoine et à la culture ! On travaille dans l'intérêt national et, dans n'importe quelle petite ville, n'importe

y a danger pour notre patrimoine et pour notre culture. je n'ai pas peur de rentrer dans mon département pour défendre l'ABF. M. le ministre disait que, lors d'un changement d'ABF, il y a quelquefois des drames ; mais il y a aussi des changements d'élus qui peuvent être destructeurs de patrimoine. On a parlé de deux prérogatives ; il y en a une dont on ne parle pas, celle de la délimitation du périmètre de protection.

Chers amis, chers collègues, les civilisations ont une durée de vie, et le grand Cioran disait que tout effort humain est voué à l'archéologie. Donc, ne détruisons pas notre patrimoine.

dans l'appréciation que l'on peut porter sur un projet de construction. Contrairement à ceux qui voient une opposition systématique ou très fréquente entre les ABF et les maires, je pense pour ma part que les ABF, à condition

que, au détour de diverses lois, on entame sans cesse davantage la capacité d'intervention des ABF. Je le sais, il peut y avoir des situations de blocage entre les élus et les ABF, mais je suis sincèrement inquiète pour notre patrimoine. Sa pérennité, la transmission de ce qui constitue l'héritage commun artistique, historique ou naturel de tous les Français doit être notre préoccupation majeure.

et l'habitat indigne, insalubre et menaçant ruine avec arrêté de péril. La vérité est que l'on ouvre la boîte de Pandore. Une fois la légitimité de l'ABF entamée, il sera plus facile de continuer à l'éroder pour d'autres types de travaux. L'avis dit « conforme » ne sera ainsi bientôt qu'un vieux souvenir, et le patrimoine disparaîtra ou tombera en ruine. Dans cet article, plusieurs autres dispositions nous posent problème. Dans le cadre du projet de décision que l'autorité compétente pourrait proposer à l'ABF pour une autorisation de travaux, la rapporteur au fond de la commission des affaires économiques a substitué un simple un simple avis consultatif à l'accord de l'ABF prévu par le projet de loi initial. Autre disposition qui nous gêne : le silence du préfet de région vaudra désormais acceptation de la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, alors que, actuellement, il vaut rejet. Cette inversion est également de nature à fragiliser la capacité d'intervention

en faisant un procès tout à fait excessif à notre position. Encore une fois, il ne s'agit ni de supprimer les ABF ni de supprimer leur avis. En outre, considérer que les maires

! Si l'on devait détruire ou considérer comme inintéressants les immeubles d'habitation insalubres ou en péril,

et aux maires pour trouver la juste voie.

ou internationaux, sur lesquels il est très difficile de communiquer. Et je comprends parfaitement que les élus aient des difficultés à comprendre que le site qui est sur leur territoire est exceptionnel et que l'on n'en trouve pas de pareil ailleurs. Par ailleurs, je veux le répéter, nous parlons de l'avis conforme des ABF,

Nous le savons, les experts désignés par les tribunaux administratifs ne sont pas toujours spécialisés dans le patrimoine ancien et ne savent donc pas toujours juger. Les rapports de ces experts- en tout cas dans la Drôme -étant très variables pour une même situation- par exemple, l'un va demander la dépose des vitres des fenêtres pour éviter les chutes de verre, tandis que l'autre va demander la démolition de l'immeuble -, l'avis conforme aide les maires, non pas pour se décharger de leurs responsabilités, mais bien pour avoir l'assurance que la décision prise est circonstanciée et éclairée. Les services municipaux n'ont généralement pas, eux non plus, de compétences en structures anciennes. Le rôle de l'ABF, par son avis conforme, permet d'apporter des solutions souvent essentielles face à une situation de péril. Je me permets de vous citer deux exemples drômois. À Valence, en 2017, rue Bouffier, l'expert conclut à la démolition totale de l'édifice.

sans solution. L'ABF est intervenu sur l'arrêté de péril en demandant l'intervention d'un ingénieur spécialiste en bâtiments médiévaux. Le nouvel arrêté de péril pris par la ville a permis de réaliser d'office les 160 000 euros de travaux nécessaires. Aujourd'hui, l'immeuble est sauvé et va être réhabilité. C'est un bijou de notre patrimoine, et l'on ne compte qu'une dizaine de bâtiments de cette qualité en France. Sans un avis conforme de l'ABF, rien n'aurait pu se faire.

Cet amendement a pour objet de maintenir l'une des prérogatives essentielles des ABF des ABF : l'initiative de délimiter un périmètre de protection. En effet, l'alinéa 1 confère cette initiative à l'autorité d'urbanisme en ne donnant à l'ABF qu'un pouvoir d'avis simple sur celle-ci. Mes chers collègues, comment peut-on

Les élus et les ABF ont tous pour objectif de protéger le patrimoine, les uns grâce à leur finalité politique et les autres de par leurs compétences techniques. Dans le cadre de l'élaboration des périmètres des abords, il paraît légitime que les élus et les ABF dialoguent.

est à M. le ministre. Par cet amendement, nous demandons le rétablissement de l'avis consultatif de l'ABF quand c'est la collectivité qui est à l'initiative de la délimitation du périmètre des abords des monuments historiques. historiques. Prévoir un accord plutôt qu'un avis de l'ABF, comme l'a proposé la commission, c'est faire perdre tout son sens à la démarche. Il s'agit plutôt d'encourager les collectivités à se saisir directement des enjeux patrimoniaux sur leur territoire, en favorisant un dialogue constructif avec l'ABF, qui restera bien évidemment associé à la définition de ces périmètres délimités. Je reviendrai d'ailleurs par la suite sur cette question de la délimitation des périmètres. Quel est l'avis de la commission

pour prévoir l'accord et non l'avis de l'ABF. En revanche, il est utile de prévoir une initiative partagée, validée par l'ABF, afin de faciliter et d'accélérer la mise en oeuvre de ces périmètres de protection.

à la lisibilité du texte. Il est ainsi mentionné de façon explicite que l'accord de la commune et de l'ABF sera nécessaire. L'initiative est ainsi élargie et le consensus est préservé. Enfin, sur l'amendement n° 782 du Gouvernement, la commission a estimé, comme je viens de le dire à l'instant, qu'il est nécessaire de préserver la validation de l'ABF sur la délimitation de ce périmètre, puisque l'initiative peut désormais être prise par la commune. L'accord double qui est prévu par les deux amendements identiques précédents permet à l'ABF et à la commune d'agir par consensus et le dialogue ainsi mis en place participe de fait à la fluidité des procédures. Donc, l'avis est défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement

autour de l'ABF comme d'autres fantasment autour du DREAL. Moi, je connais des tas d'élus qui souhaitent être accompagnés, comme l'a dit Laurent Lafon, par un protecteur,

qui feraient qu'un jour l'ABF puisse émettre un avis favorable, compte tenu de ce que je viens de dire. Personnellement, je vous invite à voter cet amendement.

Il vise à empêcher que seul un avis simple de l'ABF puisse être requis dans certains cas. D'une part, les dérogations au principe de l'avis conforme de l'ABF ne sont pas forcément justifiées au regard du faible nombre d'avis conformes défavorables rendus par les ABF, soit 6,6 %. D'autre part, ces dérogations, même limitées à seulement quatre cas, pourraient déjà se traduire par des dégradations importantes pour notre patrimoine, pourtant si précieux pour nos territoires. En effet, il ne s'agit pas de cas anodins : les dérogations pour faciliter les opérations de lutte contre l'habitat indigne, insalubre ou en péril touchent au fondement même des politiques patrimoniales telles qu'elles sont conçues depuis plus de cinquante ans, puisque l'objectif de la loi Malraux était justement d'empêcher la destruction d'immeubles très dégradés dans des zones présentant un caractère historique ou esthétique. La dérogation pour les opérations de l'ANAH pourrait être potentiellement dévastatrice : elles sont nombreuses dans les espaces protégés, y compris dans les zones qui peuvent être considérées comme des joyaux de notre pays. Je veux parler des sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, dont trente-neuf sont concernés par le plan de gestion aux termes duquel l'État français a souscrit des engagements de protection. J'ajoute que l'avis simple privera l'ABF de leviers pour entrer en négociation avec les porteurs de projet afin de trouver la solution la plus équilibrée possible compte tenu des différents intérêts en présence. Rappelons que les procédures de délimitation du périmètre intelligent des abords ou d'élaboration des documents de protection des sites patrimoniaux remarquables font systématiquement intervenir l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme pour accord, au début. Dès lors, il apparaît que, si une certaine souplesse devait être permise avec certains immeubles, c'est au moment de la délimitation du périmètre des abords et de l'élaboration du document de protection de sites patrimoniaux remarquables que le dialogue se noue naturellement entre le maire et l'ABF, occasion d'identifier lesdits immeubles qui pourraient en faire l'objet. En aucun cas il ne faut remettre en cause l'avis conforme, qui est un instrument de protection nationale de notre patrimoine sur tout le territoire.

Mais la loi a été votée à la quasi-unanimité de notre hémicycle et d'ailleurs, monsieur le ministre, vous étiez présent et j'ai apprécié les échanges que nous avons eus ensemble.

j'ai rencontré plusieurs ABF, n'en doutez pas, et j'ai dû montrer que j'étais déterminée sur les sujets dont nous avions à débattre. Cette expérience me permet d'affirmer

Il a été admirablement défendu par nos collègues. Pendant toutes ces discussions s'est manifestée une opposition entre la passion et la raison. Je citerai une phrase de l'apôtre de la raison, Descartes,

présenter l'amendement n° 67 rectifié. Si l'accès au numérique sur l'ensemble du territoire constitue une priorité, la conservation du patrimoine architectural de nos centres-villes ne doit pas être sacrifiée. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est indispensable avant d'autoriser « l'installation d'antennes relais de radiotéléphonie mobile, de leur système d'accroche au sol et de leurs locaux et installations techniques » sur des monuments historiques ou à leurs De même, l'avis conforme de l'ABF est tout autant nécessaire dans les cas de déclarations de péril et d'insalubrité, compte tenu de l'impact que peut avoir une démolition sur l'identité et le patrimoine d'une commune. Dans les sites protégés, les décisions des ABF sont généralement peu contestées- 1 % des cas, comme l'a rappelé Mme Darcos -et ne sont donc pas un obstacle au bon déroulement des procédures d'autorisation d'urbanisme. Au contraire, elles participent à la revitalisation des centres-villes et à la conservation du patrimoine bâti, vecteur du développement touristique. l'amendement n° 152. Cet amendement, comme les précédents, a pour objet de supprimer toutes les dérogations permettant de contourner les avis conformes des architectes des Bâtiments de France. Il est impensable de menacer ainsi notre patrimoine architectural. Si l'aménagement numérique de l'ensemble du territoire constitue une priorité, la richesse et la qualité de nos centres-villes historiques ne doivent pas être sacrifiées. Par conséquent, il n'est pas concevable d'autoriser l'installation d'antennes relais particulièrement peu esthétiques sur des monuments historiques ou à leurs abords sans l'accord de l'ABF. Il en est de même concernant les déclarations de péril et d'insalubrité : il n'est pas envisageable de démolir un bâtiment au caractère patrimonial avéré sans accord de l'ABF. L'argument d'efficacité économique ne tient pas. La vitalité de nos villes moyennes est indissociable de leur attractivité touristique. En préservant nos centres-villes historiques de projets peu respectueux, l'ABF joue un rôle essentiel dans leur revitalisation et dans celle des villes moyennes. Notons enfin le caractère nul et non avenu de ce dispositif. Cécile Cukierman en a parlé : les décisions des ABF ne sont quasiment pas contestées. Les élus ont bien compris l'intérêt de cet avis conforme. Ainsi, le ministère de la culture précise que sur 400 000 dossiers instruits chaque année par les ABF, moins d'une centaine ont fait l'objet d'un recours administratif. Il n'est donc ni nécessaire ni opportun de vouloir court-circuiter les ABF. La

multitude de possibilités pour installer des antennes qui ne ressemblent pas à des antennes ! J'en ai érigé une dans ma ville à côté d'un bâtiment classé, avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.

est à M. Joël Labbé. Cet amendement prévoit également de maintenir l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France en ce qui concerne l'installation d'antennes relais, au sein des périmètres relevant de sa compétence. Le développement du haut débit est un objectif qui ne doit pas mettre à mal une politique ambitieuse de protection du patrimoine. L'amendement

et l'ABF, vont dans le bon sens. Enfin, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, les maires pourront toujours s'appuyer sur l'expertise et les conseils des ABF. Ils disposeront librement et en connaissance de cause, sur ces projets nécessaires au développement économique et démographique de leur commune,

C'est la stricte réalité. Il y a patrimoine et patrimoine ... Je tenais à le dire, car nous avons voulu, avec M. le secrétaire d'État, trouver des solutions qui ne bouleversaient pas les choses, mais permettaient un équilibre par rapport à l'objectif fondamental qui est le nôtre dans ce dossier. Je remercie à cet égard Mme le rapporteur d'avoir redit que

Je sais que notre assemblée est souveraine. Malgré tout, peut-on penser que le Gouvernement et la majorité à l'Assemblée nationale aient introduit ces deux mesures dans le but manifeste d'empêcher la sauvegarde d'un patrimoine auquel nous tenons tous,

les paysages sont fabuleux, avec une diversité foisonnante, et un patrimoine qui s'enchâsse si bien dans cette exception, un patrimoine restauré et entretenu. Quelqu'un disait : « Les Français vivent au paradis et s'imaginent vivre en enfer Notre loi a protégé tout cela jusqu'à présent, elle a joué un rôle que nous ne soupçonnons peut-être pas les uns et les autres, en proposant un cadre. C'est notre responsabilité de permettre que cela continue. Il ne s'agit pas de geler quoi que ce soit, mais il faut garder la place des experts que sont les architectes des Bâtiments de France, dont les avis sont très éclairés et éclairants, comme l'a rappelé Marie-Pierre Monier. Les ABF permettent de sauver des bâtiments avec des solutions inattendues pour les non-experts que nous sommes.

En d'autres termes, ce n'est pas parce que certains ABF n'ont pas la souplesse de caractère ou la capacité de travailler sereinement avec les élus sur un projet, qu'il faut se priver de leur mission, de leur compétence et de leur avis conforme. ça ! Oui, tous les ABF ne sont pas de désagréables bloqueurs de projets, bien au contraire ! J'aimerais, ce soir, que l'on entende aussi la parole de ces élus locaux heureux avec leur formidable ABF qui les aide à ne pas mettre leur ville sous cloche,

si ! Un recours est possible grâce à la loi LCAP et au travail du Sénat qui, dans toute sa sagesse, a su allier la conviction du rôle important de l'ABF et le besoin de dialogue avec les maires et les porteurs de projets. Pourquoi remettre en cause ce qui avait été décidé ici ? Là où la communication pèche, trouvons les moyens de la médiation et du dialogue, y compris, et là je m'adresse évidemment à M. le ministre et à M. le Améliorons, mais ne brisons pas ! Les dérogations ne sont ni une solution ni la bonne approche, même pour des antennes ou l'habitat insalubre. Dans tous les cas, chacun peut trouver une solution, je vous l'assure, nous en sommes tous convaincus ici, avec son ABF dont l'avis sera conforme avec le meilleur projet, parce qu'il aura été concerté.

Mon cher collègue, nous sommes dans un champ qui est celui de l'humain, de l'appréciation. Voudriez-vous que les ABF fonctionnent de manière mathématique,

Enfin, mes chers collègues, je refuserai toujours de considérer que le pouvoir des élus et la décentralisation seraient en quelque sorte antinomiques du pouvoir de l'État républicain.

l'amendement n° 478. Cet amendement vise à revenir sur la procédure adoptée par la commission des affaires économiques, et qui consiste à prévoir une phase consultative entre le maire et l'ABF autour du projet de décision du maire. Un tel mécanisme ne paraît pas propice à accélérer les délais de procédure : quoi qu'il en soit, il faudra que le maire consulte de nouveau l'ABF, pour qu'il rende son avis conforme lors d'une phase ultérieure. procédure ne permet pas de répondre au souci, maintes fois exprimé dans cet hémicycle, que l'ABF soit plus à l'écoute des préoccupations des maires. En effet, selon ce mécanisme, c'est le maire qui soumet son projet de décision à l'ABF ; puis, ce dernier remet son avis.

s'agit d'ouvrir à l'autorité compétente, pour autoriser les travaux, la possibilité de « proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France », en amont de la procédure, afin de faciliter son accord ultérieur. Cette idée figurait du

faire l'objet d'un accord de l'ABF. La commission des affaires économiques a fait un pas en arrière en prévoyant, à la place de cet accord, un simple avis consultatif de l'ABF. Je ne comprends pas bien ce raisonnement. En effet, pour les élus,

À l'inverse, la rédaction issue des travaux de la commission est de nature à créer une culture de coopération constructive entre l'ABF et le maire pour favoriser l'autorisation des projets. Cette procédure facultative permettrait aux ABF d'indiquer en amont, aux maires, les difficultés à résoudre, afin que ces derniers ne soient pas soudainement placés face à un avis défavorable.

L'article 15 inverse la signification du silence du préfet de région ; celui-ci vaudra désormais approbation de la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux. je le rappelle, aux termes du II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, le silence du préfet vaut rejet de la décision visant à passer outre le refus d'un ABF de valider une opération susceptible de dégrader le patrimoine de la zone dans laquelle cette opération est projetée. Bref, actuellement, le silence du préfet confirme l'avis négatif de l'ABF sur un projet d'aménagement ou de travaux. L'inversion de sa signification va fragiliser le rôle des ABF, puisqu'il faudra une décision explicite du préfet pour valider son avis négatif sur un projet. Les préfets Les préfets auront-ils le temps nécessaire, dans tous les cas, pour expliquer un refus d'autorisation ? Ici encore, on complique les conditions de travail des ABF, et à quelle fin ? C'est le patrimoine qui est en jeu, et non un prétendu pouvoir qui entamerait outre mesure celui des aménageurs. Par cet amendement, nous demandons donc le maintien de la règle en vertu de laquelle le silence du préfet vaut rejet du projet de décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux.

sur l'aspect extérieur reste très limitée et dont la réalisation présente un intérêt majeur, pour le développement durable comme pour l'environnement, ainsi qu'une utilité réelle pour l'habitat.

Il appartiendrait à l'autorité compétente, à savoir, le plus souvent, le maire, d'autoriser ou non la modification demandée. Afin d'assurer un contrôle effectif des autorisations d'urbanisme, l'absence de réponse après expiration du délai d'instruction vaudrait refus.

M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement porte sur les projets modificatifs pour les permis de construire. Un projet peut être amené à évoluer raisonnablement et doit pouvoir trouver une issue dans l'instruction de l'acte réglementaire clairement définie. Si la jurisprudence définit, par exemple, la possibilité de faire évoluer un permis de construire, voire une déclaration de travaux, il apparaît nécessaire de donner plein droit à cette possibilité, tout en veillant à ce que cette demande de modification satisfasse les mêmes termes juridiques dans son examen que le projet initial et soit cohérente avec celui-ci. Dans le cas contraire, il est évident qu'une nouvelle procédure doit être engagée par le porteur du projet. Quel est l'avis de la commission

Au regard de ce constat, la création ces dernières années des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les CDPENAF, a permis d'éviter le mitage des terres agricoles et naturelles l'avis conforme rendu sur les demandes de permis de construire localisées sur ces espaces. Afin de s'assurer que les demandes et déclarations n'obèrent pas l'activité agricole et/ou les fonctions écologiques des sites concernés, il est indispensable d'accéder à des documents complémentaires tels que le statut du demandeur- agriculteur ou non -et les détails du projet renseignant sur sa viabilité technico-économique. Il est important de ne pas sous-estimer les effets du mitage qui,, réglementairement, réduisent les capacités d'épandage et le développement des filières d'élevage. Sur certains territoires restreints, ce mitage obère donc à court terme les capacités d'adaptation de l'agriculture. C'est pourquoi nous souhaitons rendre possible et même nécessaire la demande de pièces complémentaires pour les demandes et déclarations localisées sur les espaces agricoles et naturels.

Par ailleurs, si les pièces visées servent bien à la vérification du respect des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, les amendements me semblent satisfaits par le dispositif actuel.

les déclarations préalables en zones A et N. De plus, nous considérons qu'on ne peut pas laisser à l'appréciation des commissions départementales visées la composition du dossier de déclaration préalable.

Vérien, pour présenter l'amendement n° 880. Les pièces à joindre à une demande d'autorisation d'urbanisme sont limitativement énumérées par le code de l'urbanisme, ce qui interdit normalement aux services instructeurs de réclamer aux pétitionnaires des documents ne figurant pas expressément dans le code. Or, en pratique, bon nombre de pétitionnaires ont constaté que l'établissement de listes limitatives n'a pas empêché certains services instructeurs de réclamer des documents complémentaires de Cette dérive présente pour l'administration l'intérêt de prolonger le délai dont elle dispose pour examiner la demande d'autorisation, puisque le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. Le Conseil d'État, dans une décision du 9 décembre 2015, a jugé que, même illégale, une demande de pièces complémentaires prorogeait le délai d'instruction. Il convient de mettre un terme à cette dérive en prévoyant qu'une demande de pièces complémentaires illégale

mais nécessairement, pour effet de rapporter le permis de construire accordé antérieurement. Par ailleurs, le projet de loi comporte plusieurs dispositions qui faciliteront la régularisation des permis en cours d'instance.

Cet amendement vise à simplifier le droit applicable au retrait des autorisations d'urbanisme en agissant sur deux leviers. Le premier consiste à supprimer le droit de retrait de l'administration pour les déclarations préalables.

une décision expresse ou tacite de non-opposition à une déclaration préalable irrégulière peut désormais être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans un délai de trois mois suivant la date de cette décision, sans préjudice des possibilités de recours ouvertes à tout tiers lésé pendant les deux mois de l'affichage de l'autorisation. Il faut donc un mois supplémentaire pour que la décision de non-opposition soit purgée de tout recours ou retrait, ce qui retarde d'autant l'exécution des travaux prévus. Cette exception était légitimement justifiée par le fait que les demandes de déclaration préalable ne sont requises que pour les ouvrages de faible importance et pour lesquels la possibilité de retrait aurait été source de délais supplémentaires inutiles. La loi ALUR est revenue sur cette exception, sans que l'on apporte de justifications convaincantes à cette nouvelle lourdeur administrative. Il conviendrait de revenir au droit antérieur en supprimant ce droit de retrait. d'actionner consiste à aligner le délai de retrait des autorisations d'urbanisme sur celui du recours contentieux. En vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, les décisions de non-opposition à déclaration préalable et les permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacites ou explicites, peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés si celle-ci s'aperçoit de leur illégalité, dans un délai de trois mois suivant la date de ces décisions. En cas de décision explicite, la date de déclenchement du délai de retrait est celle de la signature de la décision de non-opposition ou du permis. Pour les décisions tacites, le délai de retrait court à compter de la date d'échéance du délai implicite d'acceptation. S'agissant du délai de recours contentieux à l'encontre de ces autorisations d'urbanisme, il est réglementairement fixé à deux mois. l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme prévoit que, à l'égard des tiers, ce délai court à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain de l'autorisation. Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que le titulaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable doit, avant d'être certain du caractère définitif de son autorisation, être attentif à deux risques, le retrait et le recours, soumis à deux délais distincts, dont les points de départ sont différents. Pour des raisons évidentes de simplification, il serait judicieux

parce que le délai de retrait permet aux maires, lorsqu'ils ont délivré une autorisation illégale, de faire cesser cette illégalité. Supprimer cette possibilité ou réduire le délai,

de surcroît d'être engagée. Limiter le délai de retrait des permis à deux mois priverait les maires de la possibilité de revenir sur une décision illégale. En effet, tout retrait

le délai de trois mois actuellement applicable aux autorisations d'urbanisme est déjà plus court que celui prévu dans le droit commun des actes administratifs, qui est de quatre mois. Quant à l'amendement n° 1099 de la commission,

Quel est l'avis du Gouvernement ? Cet amendement a pour objet de porter à 7 500 habitants le seuil à partir duquel les communes devront disposer d'une téléprocédure pour recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme. L'article 17 instaure une téléprocédure obligatoire pour le traitement des demandes d'autorisation à compter du 1 janvier 2022, ce qui laisse tout de même beaucoup de marge. Cette disposition a vocation à s'appliquer

La commission des affaires économiques a autorisé les collectivités à confier des missions liées à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Les auteurs de l'amendement adopté en commission font référence à la décision du tribunal administratif de Lyon du 4 mai 2017. Les conclusions du rapporteur public au tribunal administratif de Lyon rappellent qu'aucune disposition n'interdit à une collectivité d'avoir recours à un prestataire extérieur pour assurer

dans la loi la possibilité pour les collectivités de recourir à un prestataire privé afin d'assurer les missions liées à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, à condition qu'elles ne soient pas constitutives de l'instruction. Cette mission constitue pour nous un service public administratif qu'il n'est pas souhaitable

Olivier Paccaud. Par une ordonnance d'octobre 2015, l'administration a mis en place des téléservices réservés à l'accomplissement de certaines démarches administratives, notamment en matière d'urbanisme. Le législateur a ainsi mis sur un même pied l'ensemble des communes. Or nous savons tous que les petites communes n'ont pas toutes les moyens de répondre à ces exigences, en termes de matériels, mais

Avis défavorable, pour les mêmes raisons.